: « L’acétamipride, que la France n’a heureusement jamais utilisé, est pire que l’imidaclopride. Il s’agit d’un produit stable qui est donc en quelque sorte le “chlordécone de l’Hexagone”

Le scrutin est ouvert.

à l’industrie verte rendait déjà le droit moins lisible, et cette nouvelle dérogation empirerait cet état de fait. Nous demandons une stabilisation du droit relatif aux autorisations environnementales, trop fréquemment modifié.

sur des projets qui affecteront pourtant leur territoire, voire leur vie quotidienne. Les dispositifs proposés remettent en cause le dépôt d’avis par les autorités environnementales : il faudrait préciser dans la loi que ces derniers doivent être fondés sur la science… On sous entend ainsi que les décisions actuelles ne le sont pas, et qu’elles seraient dictées

simplifiant le système des ICPE ou encore en proposant de relever les seuils en deçà desquels on peut s’affranchir de l’enquête publique. Nous défendrons toujours une agriculture familiale, à taille humaine et en phase avec les attentes sociétales. Dans ce cadre, nous militons pour une agriculture soucieuse de l’environnement, qui amorce réellement sa transition agroécologique ; une agriculture respectueuse des hommes comme des animaux. Ce n’est pas en facilitant toujours davantage l’agrandissement de nos exploitations et de nos élevages, en limitant les contrôles et le dialogue démocratique, que nous serons à la hauteur des besoins et des attentes de notre société. La parole est à M. Gérard Lahellec,

Pis, en proposant d’inscrire dans la loi que les avis de l’autorité environnementale doivent être fondés sur la science, on suggère que les décisions actuelles ne le sont pas entendus posent quand même question. Enfin, cet article participe de l’instabilité du droit, donc à l’insécurité juridique, puisqu’il revient sur les dispositions de la loi Industrie verte de 2023 quant à la participation du public pour les ICPE élevage. Comme le soulignent de nombreux acteurs, en voulant « simplifier », on crée une dérogation à l’application de ce nouveau dispositif de participation du public

Dans la nuit de vendredi à samedi derniers, des activistes ont forcé l’entrée du siège social d’Evel’Up, une coopérative porcine de Bretagne. Ils ont tenté d’y mettre le feu, causant des dégâts importants, qui s’élèvent probablement à plusieurs centaines de milliers d’euros.

je propose que l’on revienne à sa rédaction d’origine. Cet amendement vise à conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement. Maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées, cette procédure s’appliquait jusqu’en 2024.

et tirées vers le bas par la loi Industrie verte. Les décrets d’application de ce texte sont entrés en application le 22 octobre dernier, et vous voulez déjà tout réécrire – évidemment, en tirant toujours vers le bas. Loin de simplifier quoi que ce soit, l’adoption d’une telle mesure complexifierait la vie de tous les acteurs, notamment les maîtres d’ouvrage, qui se sont préparés depuis un an.

C’est pourquoi, en commission, nous avons donné la possibilité au commissaire enquêteur de remplacer les deux réunions publiques obligatoires, au début et à la fin de l’enquête publique, par de simples permanences en mairie.

nous vous proposons d’aller encore un peu plus loin dans la simplification de l’enquête publique née de la loi Industrie verte en prévoyant, par cet amendement, que les réponses aux observations du public sont facultatives. Ainsi, seule la réponse à l’avis de l’autorité environnementale demeurerait obligatoire. Quant aux porteurs de projet qui souhaiteraient tout de même apporter des réponses aux remarques du public, ils pourraient procéder en une seule fois.

pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne des directives sur les

Aujourd’hui, on s’en remet à l’interprétation satellitaire, qui a montré ses imperfections. J’en veux pour preuve un exemple très concret, que j’ai déjà eu l’occasion de citer

le rapporteur propose une feuille de route pour perfectionner le fonctionnement de l’assurance récolte destinée aux prairies, sur la base d’un travail partenarial avec l’ensemble des parties. Je pense que c’est une bonne méthode.

Ils se sont rapprochés de la profession pour négocier avec elle la rédaction de cet article

un ouvrage de stockage d’eau pour une activité agricole comme d’intérêt général majeur et en inscrivant le principe de « non régression du potentiel agricole » dans le code de l’environnement. Ce faisant, il remet en cause l’ensemble de la politique sanitaire et écologique de la gestion de l’eau.

En l’absence de tout encadrement et de toute distinction entre les usages agricoles de l’eau, cet article favorise les pratiques intensives et ouvre la voie à l’accaparement des ressources par les acteurs dont les moyens financiers sont suffisants pour réaliser des ouvrages.

Cet article nous apparaît davantage comme un tract politique, visant à donner des gages à une partie des représentants du monde agricole, qu’à une réforme réfléchie de notre modèle de gestion de la ressource en eau en agriculture.

Mais une telle réforme doit faire l’objet d’un texte de loi à part entière, fondé sur la concertation de tous les acteurs, accompagné d’une étude d’impact solide et documentée, nourrie notamment de la littérature savante. À cet

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

dont le M. Premier ministre a annoncé la tenue prochainement, les dispositions relatives aux Sdage, aux Sage et à la hiérarchie des usages de l’eau.

ne me décevez pas

Cet amendement vise à supprimer l’article 6. Dans la version initiale du texte, ce dernier limitait les procédures judiciaires contre les auteurs d’infractions environnementales.

cachait à peine la volonté de proposer une réorientation des missions de l’OFB vers la prévention et l’accompagnement, au détriment d’un pouvoir de police pourtant indispensable pour protéger les milieux naturels. Voilà pourquoi nous nous étions fermement opposés à l’adoption de ce rapport. L’article 6, tel qu’il a été réécrit en commission,

texte attaque directement les outils de contrôle et de surveillance environnementale en affaiblissant le pouvoir de l’Office français de la biodiversité. Une fois de plus,

Mme la ministre.

des affaires économiques.

Le scrutin est ouvert.

d’améliorer les leviers mobilisables par les services de l’État à l’encontre des propriétaires ne prenant pas les mesures de lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine.

de limiter la dissémination de ces ravageurs, il faut prendre des mesures de lutte collective le plus tôt possible après l’identification d’un foyer. Ainsi, il faut arracher au plus vite les vignes malades et détruire les végétaux infestés.

à vous remercier.

Monsieur le président, madame la ministre,

je ne sais même pas si vous avez prononcé ces termes ! Vous vous appuyez uniquement sur des arguments économiques et de compétitivité. Vous prétendez défendre les paysans, mais en réalité vous négligez leur santé. Au sujet de l’environnement, au moins, vous êtes sincères : vous ne prétendez même pas vouloir le préserver.

On exploite les sols. On exploite les ressources. Ce modèle est tout sauf durable, et je regrette sincèrement que l’on poursuive dans cette voie.

ainsi que Mme la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, qui n’a eu de cesse de nous soutenir dans cette démarche visant à rapprocher des points de vue que l’on nous disait inconciliables.

Merci,